la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » contient quatre programmes qui relèvent de plusieurs ministères. La budgétisation proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 sur ces programmes traduit les engagements présidentiels en matière d'inclusion, de protection des personnes vulnérables et de lutte contre les inégalités pris dans le cadre de l'acte II du quinquennat. L'action du Gouvernement vise ainsi à apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. Dans cette optique, les crédits présentés dans ce projet de loi s'inscrivent en hausse de 8 % par rapport à ceux ouverts en loi de finances initiale pour 2019, soit près de 1,8 milliard d'euros de crédits supplémentaires pour mettre en oeuvre les politiques en faveur des travailleurs pauvres, des familles vulnérables, des personnes dépendantes et de celles en situation de handicap, ainsi que pour lutter contre les inégalités et violences faites aux femmes. Les principales réformes portées et financées dans le cadre du présent projet de loi de finances concernent cinq priorités. priorité, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée par le Président de la République le 13 septembre 2018 est assortie d'un budget de 8,5 milliards d'euros sur le quinquennat. stratégie est mise en oeuvre depuis 2019 et s'appuie sur de nouvelles modalités de conduite de l'action publique : la contractualisation entre l'État et les départements et la participation des personnes concernées. Le programme 304 porte l'essentiel des crédits destinés à mettre en oeuvre les engagements de cette stratégie. Des mesures importantes, emblématiques et concrètes en matière de prévention ont été lancées en 2019

-se sont engagés, ainsi que deux métropoles, Toulouse et Nantes. Les actions inscrites dans les conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi portent essentiellement sur le soutien à la parentalité, la protection maternelle et infantile, la levée des freins périphériques à l'emploi, l'inclusion numérique, l'accès à l'alimentation, la participation des personnes et la réussite éducative. Ainsi, un an après son démarrage, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présente des réalisations concrètes dans nos territoires. En 2020, 219 millions d'euros de crédits du programme 304 seront consacrés à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, dont une enveloppe de 175 millions, en hausse de 40 millions par rapport à 2019, sera consacrée à la deuxième année de contractualisation avec les départements. priorité, depuis le 1 janvier 2019, la prime d'activité est revalorisée de 90 euros au niveau du SMIC dans le cadre des mesures d'urgence économiques et sociales. Cette réforme permet d'augmenter les montants moyens de prime d'activité versés, mais également d'ouvrir le bénéfice de la prime d'activité à de nombreux foyers qui y deviennent éligibles. En un an, le nombre d'allocataires a ainsi crû de 52 %, soit 1,25 million de nouveaux bénéficiaires de la prime en 2019. Couplée à la hausse du SMIC, elle permet désormais d'offrir un gain mensuel de pouvoir d'achat atteignant jusqu'à 100 euros pour un travailleur rémunéré au SMIC.

sera étendue à compter du 1 janvier 2020 au département de La Réunion, soit 0,7 milliard d'euros de crédits supplémentaires inscrits au programme 304. Au total, la recentralisation du RSA dans ces trois territoires ultramarins concerne 127 000 personnes. quatrième priorité porte sur les politiques visant à l'autonomie des personnes en situation de handicap, dont le programme 157 est l'un des leviers au-delà de l'inclusion dans le milieu ordinaire de vie, notamment de vie professionnelle. Sur ce programme, la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) destinée à lutter contre la pauvreté subie des personnes qui se trouvent plus éloignées du marché du travail constitue un engagement présidentiel majeur. Le montant de la prestation a ainsi été porté à 860 euros par mois à compter au 1 novembre 2018 et il a été de nouveau revalorisé en novembre 2019 pour atteindre un montant de 900 euros mensuel pour une AAH à taux plein. Cette allocation bénéficie à 1,2 million de foyers. Cette mesure représente un engagement sans précédent en faveur du pouvoir d'achat des personnes éloignées du marché du travail du fait de leur handicap : plus de 2 milliards d'euros sur le quinquennat.

2020 sera l'année de concrétisation des mesures élaborées dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales lancé le 3 septembre dernier par le Premier ministre et dont les annonces ont été dévoilées lundi 25 novembre. Alors que près d'une femme meurt tous les trois jours des violences qu'elle subit, ce Grenelle sonne la mobilisation générale avec la présence d'acteurs de terrain, de professionnels, d'associations et de familles de victimes, mais également de l'ensemble du Gouvernement, notamment la garde des sceaux, Nicole Belloubet, le ministre chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie, le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, et le ministre de l'éducation nationale Au-delà des moyens financiers qui viendront en appui des actions qui seront mises en oeuvre, cette mobilisation générale vise une transformation ambitieuse des pratiques professionnelles et la mise à la disposition des acteurs d'une palette d'outils opérationnels et adaptés à la protection des victimes et de leurs enfants.

des femmes. La situation des femmes en situation de handicap est particulièrement préoccupante, puisqu'elles se retrouvent dans un état de totale dépendance face à leur conjoint en cas de violences conjugales. l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne estimait à 34 % la proportion des femmes en situation de handicap qui avaient subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire. Si 60 % des personnes voient le montant de leur allocation augmenter, tel ne sera pas le cas pour 40 % d'entre elles. La mesure que nous défendons permettra aux 250 000 bénéficiaires de l'AAH qui vivent en couple de recouvrer leur autonomie financière et de bénéficier pleinement de l'augmentation de l'AAH. Je trouve que c'est un principe que nous devons affirmer clairement et de façon solennelle par le vote d'un amendement qui rétablit les droits à l'autonomie de chacune des personnes handicapées. Quel est l'avis de la commission ? Cet

dignes aux personnes dont les ressources sont les plus faibles du fait de leur situation de handicap. Le choix qui est fait est de concentrer la solidarité nationale sur ceux qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi le calcul de l'AAH, comme comme celui des autres minima sociaux, tient compte de l'ensemble des ressources du foyer, en cohérence avec l'objectif de lutter contre la pauvreté. Pour autant, les modalités de prise en compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un bénéficiaire de l'AAH sont plus favorables que pour les autres minima sociaux, ce qui en fait une prestation quasi individualisée. Les règles de calcul de l'AAH tiennent totalement compte des besoins spécifiques de ses bénéficiaires.

la vocation de cette allocation. Vous nous dites que c'est un minima social. Je considère pour ma part qu'il s'agit d'un revenu de remplacement pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler et, par conséquent, d'obtenir un salaire. M. le

précisément identifié et justifié en prévisionnel dans le projet annuel de performance et en exécution dans le rapport annuel de performance. Ainsi, l'effort financier de l'État à l'appui de l'exercice par les départements de leurs compétences est bien inscrit en loi de finances. Le Parlement est ainsi pleinement informé du montant inscrit en PLF, puis du montant effectivement exécuté. Il ne serait pas de bonne gestion de fragmenter le budget de l'État en autant de programmes qu'il existe de dispositifs. Je pense que les membres de la commission

Pour toutes ces raisons, il semble indispensable de renforcer le réseau de nos attachés de sécurité sociale dans les principaux postes diplomatiques et consulaires à l'étranger. Je ne suis pas sûr d'avoir bien d'avoir bien mesuré le besoin de financement lié à cette action, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation actuelle, avec de moins en moins d'attachés sociaux et, partant, des coopérations de moins en moins

? Cet amendement vise à abonder les crédits du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative de 1,7 million d'euros pour créer dix postes de conseillers sociaux auprès des ambassades de France à l'étranger, afin de soutenir l'application des conventions de sécurité sociale signées avec un certain nombre d'États Je rends compte ici de l'avis de la commission des finances, qui est défavorable à l'amendement, et ce pour deux raisons : d'une part, l'augmentation de masse salariale se fait sans le plafond d'emplois correspondant ; d'autre part, le suivi des conventions de sécurité sociale n'entre pas dans le champ d'attribution des conseillers sociaux, d'après les informations communiquées par le Gouvernement.

de mon groupe. Le 7 juin 2019, la presse révélait l'affaire dite des faux steaks. En effet, dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis,

Elles ont d'elles-mêmes retiré les faux steaks. Ce faisant, elles ont eu à subir des frais importants, notamment pour faire des tests.

Le sujet est particulièrement important, bien évidemment pour les personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, mais aussi en raison de ses implications financières. Nous sommes favorables à cet amendement, ... Très bien ! ... puisque l'État s'était engagé à compenser les coûts de stockage, comme cela a été parfaitement rappelé.

Vous nous dites : « L'État a mobilisé 2 millions d'euros en autorisations d'engagement sur le programme 304, avec 500 000 euros de crédits de paiement en 2019 et 1,5 million d'euros de crédits de paiement en 2020. » Cependant, aucun de ces crédits n'est fléché dans le projet de loi de finances.

ensemble. Je vais vous indiquer très brièvement où en est la procédure. Les agissements du titulaire du marché des fournitures de steaks hachés au profit du fonds européen font l'objet désormais d'une enquête pénale à la suite des procès-verbaux établis par la DGCCRF. Cette instruction pénale permettra de déterminer les responsabilités. L'État, FranceAgriMer et les associations qui distribuent l'aide alimentaire se sont portés parties civiles afin de voir réparés les préjudices subis. De plus, une déclaration à l'Office européen de lutte antifraude a été faite.

42 % de ces enfants ont moins de six ans. J'ai le regret d'ajouter que, dans 68 % des cas, l'enfant est présent lorsque sa maman est victime de ces violences.

uniquement de l'ordre de la parole. Or il nous faut des actes. Cet amendement vise à pourvoir une ligne de crédits afin que des dispositifs d'accompagnement puissent être mis en place.

généralisons des unités d'accueil et d'écoute spécialisées à l'horizon de 2022 pour recueillir la parole de l'enfant dans de bonnes conditions et lui permettre de bénéficier d'une première prise en charge. Nous souhaitons garantir à chaque enfant victime une évaluation de ses besoins et l'accès à un parcours de soins, notamment psychologiques. parcours de soins, notamment psychologiques. La prise en compte globale de la situation de ces enfants implique la mobilisation de l'ensemble des ministères et de plusieurs missions budgétaires : cohésion sociale, santé, justice, éducation nationale. Aussi, réduire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes à un programme doté de 1 million d'euros pour des actions relevant du seul champ de la cohésion sociale

L'ouverture du 119 au-delà des heures habituelles ne va pas répondre à la question de la prise en charge des enfants orphelins de mère et dont le père est condamné pour crime. Le Premier ministre a annoncé qu'en cas de féminicide le père perdrait l'autorité parentale. Il s'agit donc d'enfants qui deviendront des pupilles, très probablement. Ces enfants-là ont besoin d'un suivi particulier. Or vous n'avez rien prévu de tel. Quand bien

C'est un engagement réel, ample, profond et sincère que le pays attend. Les dizaines de milliers de femmes mobilisées la semaine dernière devraient vous faire entendre raison. La parole est

Alors que ces crédits sont en baisse d'un demi-million d'euros entre la loi de finances pour 2019 et le projet de loi de finances pour 2020 et que les associations connaissent un afflux sans précédent de demandes à la suite du mouvement #MeToo, cet amendement tend à dégager des crédits supplémentaires pour financer les subventions aux associations, les dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violence, c'est-à-dire des places d'accueil, les référents départementaux, ou encore la plateforme téléphonique 3919. Cet amendement a pour objet de conduire le Gouvernement à apporter des moyens nouveaux pour ces actions et, plus largement, hors du périmètre de cette mission, pour financer les mesures annoncées dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. En effet, à ce jour, aucune mesure n'est clairement financée.

est à M. Julien Bargeton. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Patricia Schillinger. La précarité liée aux règles était jusque récemment un sujet assez peu connu et peu abordé en France. Faute de moyens, beaucoup de femmes dans notre pays se retrouvent dans l'impossibilité de se procurer

ainsi que les établissements d'enseignement, puisque certaines jeunes filles et jeunes femmes scolarisées ne se rendent pas en cours à l'école ou à l'université pendant leurs règles faute d'accès suffisant à des protections périodiques. Ce rapport a été bien accueilli par les acteurs de la solidarité, de même que par l'Assemblée des départements de France, puisque certaines collectivités s'engagent également dans ce chantier face à un fléau tant social que sanitaire. Plus techniquement, le dispositif allège de 1 million d'euros les crédits

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à abonder les crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à hauteur de 700 000 euros, et ceux du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », de 300 000 euros, afin de mener une expérimentation de libre distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du public, notamment les plus vulnérables, comme les centres d'hébergement d'urgence, les associations caritatives et les lieux d'enfermement. La commission a émis un avis défavorable.

propose une expérimentation. Le Gouvernement est sensible à cette proposition, qui est à l'étude sur la base des chiffrages que Mme Schillinger a établis. En parallèle, la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale s'est mobilisée pour produire un rapport complémentaire sur les problématiques multidimensionnelles qui entourent les règles et les produits d'hygiène.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à augmenter de 800 000 euros l'enveloppe dédiée à l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle des personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution, qui est passée de près de 2 millions d'euros en 2019 à 1,2 million d'euros en 2020. Alors que 40 000 personnes seraient victimes d'exploitation sexuelle en France, l'effort en faveur de cette politique mérite d'être soutenu. La forte réduction de l'enveloppe qui lui est consacrée constitue un très mauvais signal.

En effet, alors que le nombre de bénéficiaires de cette prestation ne cesse de diminuer du fait de conditions très restrictives, les crédits demandés s'élèvent à 4,5 millions d'euros pour 2020, contre 1,7 million d'euros en loi de finances initiale pour 2019.

Il y a deux ans, Éric Bocquet et moi-même nous étonnions déjà de la sous-consommation de ces crédits. On nous avait alors expliqué qu'il fallait un certain temps pour mettre en place les commissions départementales qui décident de les attribuer dans le cadre des programmes de sortie de la prostitution.

La réduction, entre 2019 et 2020, des crédits de l'AFIS inscrits en loi de finances résulte d'une montée en charge plus modérée qu'initialement prévu du nombre de bénéficiaires de cette prestation réglementaire.

Vous ne prenez aucun engagement en faveur de l'application de ce texte et du parcours de sortie de la prostitution. J'en veux pour preuve que vous n'en parlez jamais. jamais. Quand vous parlez des violences faites aux femmes, faites aux personnes, jamais vous ne citez la prostitution parmi ces violences. Jamais vous ne parlez de la traite des êtres humains : cela n'existe pas dans le vocabulaire et le paysage mental de ce gouvernement.

leurs premières parties. Quand on vote l'impôt, en général, il est appliqué immédiatement. Quant aux autres lois, il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller en faire la promotion, y compris auprès des fonctionnaires.

? Le présent amendement porte sur l'article 78, qui réforme l'aide à la réinsertion familiale et sociale. Il vise à clarifier les conditions d'éligibilité au dispositif. L'avis de la commission est favorable, car cet amendement cet amendement clarifie utilement certaines dispositions de cet article relatives à cette nouvelle aide à la vie familiale et sociale, en supprimant la condition d'hébergement dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale pour le maintien de l'aide et en réintroduisant les dispositions prévoyant une revalorisation annuelle de l'aide.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le budget de l'enseignement supérieur pour 2020 s'inscrit dans la trajectoire dessinée par la loi de finances pour 2019, avec une nouvelle hausse des crédits, de l'ordre de 242 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 1,5 % par rapport à 2019.

Dans le détail, le budget pour 2020 affiche une hausse de 159 millions d'euros des crédits dédiés aux formations supérieures et à la recherche. Bien évidemment, madame la ministre, je ne peux que saluer cet effort budgétaire manifeste en faveur du plan Étudiants, de la réforme des études de santé et de l'expérimentation du dialogue stratégique et de gestion. Je voudrais néanmoins vous faire part de quelques réserves quant à la présentation que vous nous faites de ces augmentations de crédits. J'ai pu constater au cours de mes travaux qu'une grande partie des moyens présentés comme nouveaux correspondaient en réalité au financement de dépenses obligatoires ou à la prolongation, en année pleine, de mesures décidées en 2019. près du quart de cette enveloppe de 159 millions d'euros a vocation à compenser le coût du dispositif « Parcours professionnels, carrières et rémunérations Par ailleurs, alors que vous avez annoncé la fin de la compensation systématique du GVT, une partie des 50 millions d'euros dédiés au dialogue stratégique et de gestion devrait être mobilisée pour octroyer à certains établissements, au cas par cas, une compensation partielle ou totale. Pourriez-vous me dire quel montant sera finalement dédié à la compensation du GVT ? Si je soutiens pleinement l'expérimentation de ce dialogue de ce dialogue stratégique, je remarque que,, seuls 15 millions d'euros seront consacrés au financement des projets stratégiques de 80 établissements,

dont 30 millions d'euros au titre de l'extension en année pleine des mesures attribuées pour la rentrée de 2019. J'adhère pleinement aux mesures de ce plan, qui accorde une grande importance à l'orientation des élèves, afin notamment de réduire l'échec en licence.

sans pour autant bénéficier d'un accompagnement financier adéquat de l'État. En 2019, les établissements privés ont accueilli 9 500 étudiants de plus que l'année dernière, ce qui correspond à une hausse de 9 % de leurs effectifs. Pourtant, tandis tandis que l'université voit sa dotation progresser de plusieurs dizaines de millions d'euros en 2020, les Eespig, c'est-à-dire les établissements qui ont contractualisé avec votre ne bénéficieront que de 3 millions d'euros supplémentaires pour accompagner cette hausse d'effectifs. En 2020, les Eespig représenteront 4 % des étudiants de l'enseignement supérieur, mais ne percevront que 0,6 % des crédits du programme 150. Mécaniquement, le montant moyen de la subvention de l'État par étudiant, qui a diminué de 46 % entre 2009 et 2019, va continuer de chuter.

L'enseignement supérieur est confronté à un deuxième défi, à savoir la diversification de ses ressources. Je suis extrêmement inquiet des conséquences que pourrait avoir la réforme du mécénat sur le financement de l'enseignement supérieur, des grandes écoles comme des universités. Il me semble pour le moins paradoxal que l'État ne cesse d'inciter les établissements à développer et à diversifier leurs ressources propres et que, en parallèle, il diminue sans vergogne les dispositifs encourageant les entreprises à financer l'enseignement supérieur.

En 2020, les crédits du programme 231 augmenteront de 66,4 millions d'euros par rapport à 2019, ce qui rompt avec la stabilité observée jusqu'à présent. Je note ainsi que le montant inscrit au titre des bourses sur critères sociaux progresse de 46 millions d'euros, en raison, d'une part, de la revalorisation de ces bourses et, d'autre part, de l'augmentation prévisionnelle du nombre de bénéficiaires. Cette hausse constitue bien évidemment un signal positif, mais elle ne saurait constituer une réponse à la crise étudiante actuelle. J'identifie pour ma part deux sujets majeurs

Monsieur le président,

Il va sans dire que ce texte est attendu : les travaux préparatoires à son élaboration ont suscité de grands espoirs chez nos chercheurs, qui demeurent suspendus aux annonces qui pourraient être faites dans les mois à venir. La recherche étant une dépense d'avenir par excellence, s'inscrivant plus que toute autre dans le temps long, je me félicite que le Gouvernement s'attelle à l'élaboration d'une loi pluriannuelle. Néanmoins, madame la ministre, vous le savez, la tâche est immense et les défis ne manquent pas attractivité des carrières scientifiques, soutien à la recherche publique, amélioration des performances à l'échelle européenne ... J'espère vivement que le texte que vous nous présenterez sera à la hauteur de ces enjeux et portera une véritable ambition pour la France. Dans ce contexte, le projet de budget pour 2020 est un budget d'attente et de transition : les crédits demandés pour 2020 sont conformes à la programmation pluriannuelle et ne rompent pas avec les grands équilibres budgétaires définis jusqu'à présent.

de 428 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 292 millions d'euros en crédits de paiement. En dépit d'un contexte budgétaire contraint, ces hausses de crédits traduisent concrètement la priorité accordée par le Gouvernement à la recherche et méritent donc

Depuis 2018, les crédits alloués à ce domaine d'excellence de la recherche française ont progressé de plus d'un demi-milliard d'euros, preuve s'il en est de l'importance stratégique de ce secteur, nous en convenons. effort budgétaire devrait garantir, en 2020, l'apurement définitif de la dette française auprès de l'Agence spatiale européenne, ce qui mettra fin à une situation difficilement compatible avec nos ambitions.

en 2020. Ces efforts sont encourageants et devraient enfin permettre à l'ANR de renouer avec un taux de succès acceptable lors des appels à projets, de nature à moins décourager nos chercheurs de candidater.

J'ai déjà eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, le financement de ces installations demeure particulièrement opaque et illisible, alors même que l'ampleur des investissements consentis, souvent sur plusieurs années, nécessiterait un suivi étroit. Madame la ministre, j'attends de pied ferme les pistes d'amélioration qui seront proposées à cet égard dans le projet de loi de programmation. De manière générale, je regrette que le financement de la recherche soit de plus en plus éclaté. Le plan Intelligence artificielle, qui doit bénéficier de 1,5 milliard d'euros sur cinq ans, me semble particulièrement emblématique de cette dispersion des crédits. supérieur » participera à hauteur de 358 millions d'euros sur cinq ans, mais les circuits de financement retenus sont extrêmement complexes et font intervenir une multitude de structures programmes d'investissements d'avenir, le Fonds pour l'innovation et l'industrie, les missions budgétaires. Vous en conviendrez, madame la ministre, cette situation entrave considérablement le suivi et le contrôle parlementaire. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. reprises. Quatrième et dernier point : la situation des organismes de recherche. Vous le savez, au cours des trois dernières années, la masse salariale de ces organismes n'a cessé d'augmenter, en raison de la relance de la politique salariale, dont le coût n'est que partiellement compensé par l'État. Pour absorber cette hausse, la plupart des opérateurs en sont réduits à rogner sur leurs effectifs, ce qui entraîne une sous-exécution inquiétante des plafonds d'emplois. Dans ce contexte, je regrette vivement qu'il soit question d'un taux de mise en réserve de 4 %. Madame la ministre, pouvez-vous me confirmer l'application d'un tel taux en 2020 ? Le cas échéant, vous le savez, les attentes à l'égard du projet de loi de programmation n'en seront que plus grandes. Je me félicite cependant que la plupart des impasses budgétaires identifiées en 2019 aient été résolues. Je pense notamment au financement de la construction du réacteur de recherche Jules Horowitz, qui a été clarifié en cours d'année. Avant de conclure, j'évoquerai rapidement le crédit d'impôt recherche. Les travaux les plus récents sur le sujet, menés en 2019 par la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation, ont conclu à un effet multiplicateur supérieur à 1 du CIR sur les dépenses de recherche des entreprises. Ces résultats me confortent dans ma conviction profonde, à savoir que le CIR constitue une aide à l'innovation absolument déterminante et qu'il doit être préservé pour soutenir l'effort de recherche dans notre pays.

ce projet de budget marque un nouvel effort en faveur de la recherche. Cet effort porte en particulier sur la politique spatiale et les lanceurs, sur lesquels notre commission a récemment publié un rapport, conjointement avec la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées,

dans l'attente, certainement, du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. L'enjeu est de taille : notre effort en matière de recherche stagne depuis les années 1990 autour de 2,2 % du PIB. Nous dépensons deux fois moins que l'Allemagne en valeur dans la R&D. Nos politiques de recherche et d'innovation sont de plus en plus illisibles. Nous multiplions les instances et les circuits financiers. Nous ne sommes pas à la hauteur Il faut cependant saluer la pugnacité de nos chercheurs, qui parviennent à maintenir la France au meilleur niveau malgré ce manque de moyens. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la cohérence entre le discours et les actes du Gouvernement.

ailleurs également défendu, sous une autre forme, par certains de nos collègues. C'est aussi le cas s'agissant des pôles de compétitivité, qui restent au milieu du gué, ballottés entre l'État et les régions, alors que le financement des projets de recherche partenariale qu'ils labellisent diminue et devient moins lisible pour les parlementaires. Madame la ministre, ces sujets relèvent du ministère de l'économie, mais je compte sur vous pour faire passer le message. Enfin, nous sommes inquiets s'agissant des moyens des organismes de recherche et de l'Agence nationale de la recherche. Le taux de mise en réserve des crédits n'est toujours pas arrêté ; or il détermine l'ampleur des moyens véritablement mis à leur disposition et la crédibilité des informations transmises au Parlement- je pense notamment aux 30 millions d'euros de hausse des crédits d'intervention de l'ANR. Pour les organismes de recherche, le glissement vieillesse-technicité fait du personnel la variable d'ajustement

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme les années précédentes, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie pour avis des crédits du programme 190 de la mission « Recherche et enseignement supérieur En 2020, les crédits de ce programme représenteront 1,79 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1,77 milliard en crédits de paiement, soit une légère augmentation par rapport à 2019. de la mission en commission, nous nous sommes félicités de cette augmentation, même si elle reste modeste, au regard des défis à relever. À l'heure de l'accélération de la transition écologique, et alors que le Parlement vient d'examiner ou d'adopter des textes aux objectifs ambitieux comme la loi d'orientation des mobilités, la loi relative à l'énergie et au climat et, plus récemment, le projet de loi relatif à la le soutien à la recherche en matière de développement durable est déterminant et contribue au rayonnement de notre pays à l'échelon international. Nous avons toutefois regretté certaines évolutions contrastées tandis que les crédits destinés à la recherche sur l'énergie nucléaire augmentent sensiblement, les crédits destinés à la recherche dans les nouvelles technologies de l'énergie baisseront une nouvelle fois, de 2 millions d'euros.

Pourtant, depuis dix ans désormais, l'IFPEN connaît une baisse quasi constante de sa dotation. Même si cette baisse est partiellement compensée par ses ressources propres,

tout d'abord le CEA, qui, outre ses activités historiques sur l'énergie nucléaire, travaille au développement des nouvelles technologies de l'énergie. À ce propos, on ne peut que se féliciter de son projet de plateformes régionales de transfert de technologie, implantées dans six régions, qui

Enfin, je souligne les actions de recherche de l'Ineris dans le domaine des risques industriels. Ces programmes consolident son expertise déjà reconnue et dont l'utilité a été récemment démontrée lors de la gestion de l'incendie de l'usine Lubrizol. C'est pourquoi il nous semble plus que justifié de sauvegarder durablement ses ressources. Madame la ministre, notre commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits du programme.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne serai pas très originale en vous disant que 2020 sera une année charnière pour la recherche. Ce projet de budget en est l'expression.

Cet effort budgétaire, principalement porté sur la recherche spatiale, est bien sûr positif et louable. Toutefois, il n'est pas de nature à enclencher une véritable dynamique permettant de rassurer les esprits. Les attentes envers le futur projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche n'en seront que plus fortes. La stabilisation de la dotation du programme 172, qui finance les principaux opérateurs de recherche, est particulièrement révélatrice de ce contexte attentiste, générateur d'inquiétudes, voire de colère. Les organismes de recherche sont confrontés depuis plusieurs années à de graves problématiques financières, auxquelles le projet de loi de programmation devra répondre. J'en citerai trois principales. J'évoquerai tout d'abord le taux de réserve de précaution. Actuellement de 3 %, il serait porté à 4 % l'année prochaine. La confirmation de ce relèvement serait un très mauvais signal envoyé aux acteurs de la recherche, qui dénoncent les conséquences délétères de cette réserve en termes de marge de manoeuvre et de visibilité financières. le glissement vieillesse-technicité. Son financement n'est plus pris en compte depuis plusieurs années dans la subvention pour charges de service public des opérateurs de recherche, qui doivent donc l'autofinancer. Cette situation les oblige à réduire régulièrement leurs effectifs afin de contenir leur masse salariale. les modalités de financement. Le développement du financement sur projets, qui présente de nombreux atouts, ne doit pas conduire à un effet d'éviction sur le financement à travers les dotations « de base », lesquelles ne peuvent plus continuer à être absorbées par une masse salariale grandissante. La marche financière est donc haute, et le projet de budget pour 2020 ne permettra pas véritablement de l'abaisser.

Je ne peux que souscrire aux propos tenus par le Président de la République, qui, à l'occasion des quatre-vingts ans du CNRS mardi soir dernier, a rappelé « la nécessité d'un investissement dans la recherche publique, car c'est un choix de souveraineté Un autre dossier majeur est, lui aussi, toujours en attente de réponses : la valorisation du statut des chercheurs. Le constat est connu et partagé : une rémunération en décrochage par rapport aux standards internationaux et au sein même de la fonction publique française ; un recrutement particulièrement tardif une perte d'attractivité du métier et de la carrière ; une progression de l'emploi contractuel et une systématisation du recours aux vacataires. Le sujet ne se résume pas à une question financière, c'est aussi un devoir moral : il est urgent de renouer le pacte de la Nation avec ses chercheurs Vous l'aurez compris, les attentes sont si fortes que le projet de loi de programmation devra être à la hauteur, au risque sinon d'une rupture encore plus profonde, et peut-être même irrémédiable, avec le monde de la recherche, mais je crois comprendre, madame la ministre, que telle est l'ambition du Gouvernement. Sous les réserves que je viens d'émettre, et en raison de l'augmentation globale du budget, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le budget de l'enseignement supérieur proposé pour 2020 poursuit la trajectoire ascendante dessinée par la loi de finances pour 2019 2019 : les crédits des programmes 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » et 231 « Vie étudiante » connaissent une augmentation de 1,5 %, ce qui représente 242 millions d'euros supplémentaires.

défi démographique. Sous l'effet d'une croissance soutenue des effectifs, la dépense publique moyenne par étudiant suit une tendance à la baisse depuis 2010. défi de la masse salariale. Madame la ministre, vous avez récemment annoncé aux établissements que le financement systématique du glissement vieillesse-technicité ne sera plus assuré.

défi patrimonial. De nombreuses universités sont confrontées à la vétusté de leurs installations et doivent envisager des projets de rénovation importants. Or elles manquent toujours de leviers financiers pour réaliser des travaux que l'on sait très coûteux. Aussi, sans un changement d'échelle dans l'investissement public consacré à l'enseignement supérieur, ces défis ne pourront être relevés. Le secteur se trouve d'autant plus déstabilisé que la récente décision du Conseil constitutionnel sur les droits d'inscription ouvre une inquiétante période d'insécurité juridique pour les établissements, en particulier les grandes écoles. L'emploi de l'adjectif « modique » laisse en effet la place à toute une gamme d'interprétations, dans l'attente de l'analyse du Conseil d'État. J'estime, pour ma part, que les droits d'inscription sont un réel levier de financement qui mérite d'être activé, dès lors qu'il est tenu compte, bien évidemment, des capacités financières des étudiants. Un autre mode de financement propre me paraît devoir être encouragé : le mécénat, qui a déjà été évoqué. Encore insuffisamment développé en France, en comparaison d'autres pays, il est néanmoins en plein essor. Les trois quarts de nos universités se sont dotées d'une fondation, chacune percevant, en moyenne, 630 000 euros annuels. Les fonds récoltés proviennent à 87 % d'entreprises généralement implantées sur le même territoire.

C'est pourquoi je me réjouis que le Sénat, sur l'initiative de sa commission des finances et de sa commission de la culture, propose de revenir sur cette disposition, dont les effets délétères sont assurés. Sous ces réserves, et en raison de l'augmentation globale du budget, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » pour 2020.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous évoquons ce jour les crédits alloués à la mission « Recherche et enseignement supérieur », qui sont en progression d'un demi-milliard d'euros, ce qui est significatif,

de s'orienter vers « un investissement, par choix de souveraineté, et de profondes réformes ! » L'effort budgétaire consenti dans le volet « Enseignement supérieur », de l'ordre de 242 millions d'euros, servira à la revalorisation des carrières de professeurs, à l'expérimentation du dialogue stratégique et de gestion avec les universités,

et une prime spécifiques, que nous considérons comme stratégiques pour la qualité de notre enseignement universitaire. La progression des crédits permettra également d'accompagner les universités qui devront préparer la réforme des études de santé au premier semestre prochain, pour une mise en oeuvre effective prévue à la rentrée de 2020 : 6 millions d'euros sont ainsi prévus pour la réforme, auxquels s'ajouteront 11 millions d'euros débloqués en fonction des projets présentés par les établissements. restent en suspens, touchant notamment à l'accompagnement stratégique et budgétaire de la réforme. Ainsi, la variation des contenus de la « mineure santé » d'une université à l'autre doit pouvoir être maîtrisée, afin de prévenir toute inégalité dans la qualité de l'enseignement. De même, la visibilité des universités sur la répartition de l'enveloppe de 11 millions d'euros doit être améliorée, pour qu'elles aient connaissance des moyens exacts dont elles disposeront pour mettre en oeuvre la réforme à la rentrée

la conférence des doyens d'université attendait plus de moyens, condition de son appui nécessaire à la mise en oeuvre de la réforme des études de santé. Notre appréciation des crédits consacrés à la vie étudiante peut difficilement être détachée de la question de la précarité des étudiants.

Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 66 % des étudiants non pauvres bénéficient d'aides publiques, contre seulement 49 % des étudiants pauvres. L'ajustement des soutiens aux besoins réels est peut-être le véritable enjeu pour lutter contre la précarité étudiante en restreignant le nombre des bénéficiaires pour augmenter le montant Au total, ce budget pour l'enseignement supérieur nous paraît satisfaisant, même si, gardons-le à l'esprit, il constitue, comme celui de la recherche, un investissement de long terme aux puissants effets de levier. Nous pouvons et devons aller plus loin pour garder notre rang dans la compétition internationale. Si ce budget ne marque pas réellement de rupture majeure par rapport aux années précédentes, nous sommes surtout dans l'attente de la présentation du projet de loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Attendu dans le courant de l'année prochaine, ce texte devrait amorcer de plus profondes évolutions. Cette année encore, le budget de la recherche est difficilement lisible, en raison de l'éclatement du financement de la recherche dans les différents programmes d'investissements d'avenir, mais aussi dans le Fonds pour l'innovation et l'industrie. Sur le volet recherche, une hausse substantielle, de 428 millions d'euros, soutiendra les politiques d'attractivité des carrières scientifiques, le renforcement du plan Intelligence artificielle, le développement de la politique spatiale et le soutien à la création de l'Inrae au 1 janvier

pluriannuelle de la recherche à la mi-février, ce qui nous permettra, selon le voeu du président du CNRS, « de lutter à armes égales avec nos concurrents internationaux ». La parole Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chaque année, l'examen du projet de loi de finances est un grand moment de « vérité des prix

tant nos prédécesseurs ont usé et abusé de projets de loi de finances rectificative monstrueux, véritables « lois de finances qui n'osaient dire leur nom ; abusé, aussi, de niveaux surréels de mises en réserve, associés à un usage systématisé des décrets d'avance en cours d'exercice. Au fil du temps, le vrai moment de vérité des prix des politiques publiques est devenu la loi de règlement, et non le projet de loi de finances de l'année, certes âprement discuté par le Parlement, mais sournoisement révisé et reformaté en cours de route par les gouvernements qui nous ont précédés.

». La raison en est simple : cette mission est l'une de celles qui, jusqu'en 2017, ont été le plus systématiquement rognées en cours d'exercice par des avalanches de décrets d'avance et de gels de crédits. Entre les grands discours ambitieux tenus pendant plus d'une décennie et la mise en oeuvre effective des moyens, rarement le décalage n'aura été si grand. Le caractère erratique, souvent aussi très malthusien, de la dépense publique dans des domaines d'investissement stratégiques comme l'enseignement supérieur et la recherche aura eu, sur la durée, plus encore qu'ailleurs, des effets dramatiques sur le dynamisme et l'avenir de notre économie. Dans le domaine de la recherche, en particulier, la sous-budgétisation et l'absence de prévisibilité à moyen et long terme des engagements de l'État ont souvent conduit à déstabiliser un secteur hautement concurrencé et largement contribué à alimenter la crise de confiance de la communauté communauté scientifique à l'égard de l'État. Car il ne suffit pas de se doter de moyens budgétaires substantiels chaque année. Encore faut-il définir une véritable trajectoire pluriannuelle dans ce domaine et s'y tenir, en dépit des aléas

Il est bon de rappeler que le budget du ministère était resté tristement stable de 2012 à 2016, malgré de beaux discours d'intention, des discours ... Bien sûr, tout cela peut être jugé encore insuffisant, notamment au regard de l'état de délabrement de l'université et de la recherche universitaire dont nous héritons. Mais les moyens insufflés sont tout sauf de la monnaie de singe, car nous nous faisons un honneur, depuis deux ans, de ne pas recourir aux sempiternels décrets d'avance ou aux massifs gels de crédits. Au reste, nos ambitions ne s'arrêtent évidemment pas

Horizon Europe, le plus important programme de recherche publique au monde, doté d'environ 100 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Cet investissement massif et cette synergie entre budget national et budget européen sont absolument nécessaires si nous ne voulons pas que notre pays et notre continent soient définitivement dépassés dans la rude compétition qui nous oppose aux États-Unis, à la Chine et aux autres puissances émergentes.

pendant plusieurs années omis de s'acquitter de la contribution de la France ... Avec l'augmentation de 213 millions d'euros des crédits du programme 193, notre pays aura presque achevé d'apurer la dette contractée. comme dans bien des domaines, le Gouvernement, loin de la démagogie et des faux-semblants de ses prédécesseurs, s'honore de respecter les engagements pris par d'autres, qui ne les avaient pas tenus. Lors de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, qui s'est achevée hier à Séville,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à cette même tribune, l'an passé, j'avais appelé votre vigilance sur les prodromes flagrants d'un décrochage de l'enseignement supérieur et de la science français. Les groupes de travail chargés de la réflexion préparatoire à l'élaboration de la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche viennent de confirmer ces inquiétudes et dressent un bilan partagé de cet état préoccupant.

depuis bientôt dix ans, les dépenses de recherche croissent moins vite que le produit intérieur brut. Elles représentaient encore 2,28 % du PIB en 2014 ; 2,19 %. L'effort budgétaire de l'État dans ce domaine est médiocre et bien inférieur à celui de nos voisins européens. Quant aux sommes investies par les entreprises privées

la faiblesse chronique des investissements a des conséquences funestes pour l'emploi scientifique et l'attrait des étudiants pour les carrières scientifiques. La France est ainsi l'un des rares pays d'Europe dont le nombre de doctorants est en baisse constante. Cette régression doit être rapportée à la chute drastique des recrutements par les opérateurs publics

Dans ces conditions, c'est la validité scientifique même des concours qui est fragilisée. En effet, par découragement, de nombreux jeunes chercheurs quittent notre pays. Cette fuite des cerveaux est un symptôme de plus du déclin de la science française.

il s'inscrit dans un cadre qui a imposé à l'enseignement supérieur et à la recherche une progression budgétaire inférieure à la moyenne des crédits de l'État. Au-delà des effets d'annonce et de la promotion de mesures nouvelles, plusieurs déficits structurels vont nécessairement continuer, en 2020, d'affaiblir la situation économique des opérateurs de la mission. Ainsi, l'absence de compensation du glissement vieillesse-technicité oblige les opérateurs à réduire leur masse salariale. Pour les universités, cette perte conduit au gel de plus de 1 200 emplois. Je regrette vivement, avec nos rapporteurs, que le Gouvernement demande au Parlement de se prononcer sur des objectifs qu'il sait inaccessibles. De la même façon, dans un contexte de hausse de la démographie estudiantine, la quasi-stabilité des moyens alloués aux universités aboutit à une baisse du budget moyen par étudiant. Ce ratio est en diminution de près de 1 point tous les ans depuis 2010. Pour 2018, il a été estimé à 11 470 euros, son plus bas niveau depuis 2008.

le Gouvernement veut aller plus vite : il a décidé d'augmenter le niveau de la réserve de précaution de 3 % à 4 %. Le précédent de la loi de finances rectificative, adoptée cette semaine, révèle que, pour l'enseignement supérieur et la recherche, les crédits gelés en début de gestion budgétaire sont intégralement annulés à la fin de l'année. Mes chers collègues, nous débattons donc d'un budget qui sera encore plus diminué l'année prochaine par ces annulations. À tout cela, il faut ajouter le refus du Gouvernement d'anticiper les conclusions de la récente et inédite décision du Conseil constitutionnel. Grâce à votre décret sur les droits d'inscription différenciés, les Sages ont considéré que l'enseignement supérieur était constitutif du service public de l'éducation nationale et que le principe de gratuité s'y appliquait. Le Conseil constitutionnel admet toutefois qu'il est loisible aux établissements de percevoir des droits d'inscription, à la condition expresse qu'ils restent modiques par rapport aux capacités contributives des étudiants. Il n'est point besoin d'attendre l'interprétation que donnera le Conseil d'État de cette décision pour supposer que celle-ci ouvre des voies de recours à tous les étudiants qui considèrent leurs frais d'inscription comme disproportionnés. Ces possibles contentieux risquent de priver de nombreux établissements de ressources importantes. En théorie, votre projet de budget paraît quasi stable ; en pratique, il risque de s'avérer encore plus déficient que l'an passé. À tout le moins, il n'est pas la manifestation budgétaire d'une priorité politique en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au reste, vous en avez parfaitement conscience, puisqu'il nous est demandé d'attendre le début de l'année prochaine pour connaître des ambitions du Président de la République en ces matières. nous débattons donc d'un projet de budget des affaires courantes, les annonces décisives étant réservées à un autre auditoire. Il en va du budget de la recherche comme de celui de la sécurité sociale : l'essentiel n'est pas destiné à cet hémicycle ... Nous voterons contre ces crédits

de la vie étudiante et de la recherche dans l'ensemble des domaines couverts par l'État. Contrairement à l'orateur précédent, mon groupe salue l'engagement du Gouvernement en faveur de cette mission stratégique pour l'avenir de notre économie. chercheurs et étudiants bénéficieront l'année prochaine de 534 millions d'euros de crédits supplémentaires, le budget atteignant 28,68 milliards d'euros, soit 10 % des dépenses pilotables. Il faut admettre que la France demeure bien en deçà de l'objectif de Lisbonne- 3 % du PIB investi dans la R&D -, contrairement à l'Allemagne et aux pays scandinaves. Or notre compétitivité par rapport aux puissances étrangères et aux grandes entreprises technologiques dépend directement de l'excellence de nos formations, de l'engagement de la France dans les recherches de pointe et de notre capacité à attirer et garder les jeunes talents. La France dispose de nombreux atouts, mais les opportunités ouvertes par les innovations technologiques des vingt dernières années sont immenses. Nous ne pouvons pas nous résigner à être seulement utilisateurs de ces technologies. Le financement de cette mission est une question de souveraineté nationale. À travers le financement de la recherche et l'excellence de nos formations, il s'agit de nous positionner en acteurs du changement et de réunir aujourd'hui les conditions nécessaires à l'émergence des solutions de demain pour répondre aux défis du siècle. Bien sûr, il s'agit là d'un budget de transition, dans l'attente de l'examen par le Parlement du projet de loi de programmation de la recherche. Cette réforme, très attendue par la communauté scientifique, devrait permettre de donner davantage de visibilité aux laboratoires et de renforcer l'attractivité des carrières. Le premier programme de cette mission, doté de 13,6 milliards d'euros, est consacré aux formations supérieures et à la recherche universitaire. Ses crédits permettront notamment la poursuite du plan Étudiants et la réforme des études de santé pour favoriser les passerelles entre formations et diversifier les profils. Le programme « Vie étudiante » bénéficiera l'année prochaine de 175 millions d'euros supplémentaires, pour atteindre un montant de 2,7 milliards d'euros. Le Gouvernement a fait le choix de renforcer les moyens consacrés aux bourses sur critères sociaux, à hauteur de 46 millions d'euros, sans revaloriser l'aide au mérite, dont le montant a été divisé par deux en 2015. Le manque de places en résidences universitaires cause un véritable problème de précarité pour les étudiants, qui dépensent en moyenne 70 % de leur budget dans leur loyer. Nous devons réagir pour garantir à chaque étudiant des conditions de vie décentes et faciliter la mobilisation des aides d'urgence. En matière de recherche, les financements permettront de développer le plan Intelligence artificielle au sein du programme 172, d'accompagner la création du nouvel Inrae, consacré à l'agronomie et aux sciences de l'environnement, et d'améliorer l'attractivité des carrières scientifiques au sein du CNRS et de l'Institut national de recherche en sciences du numérique. Comme l'a fait le président Claude Malhuret en commission, j'appelle l'attention du Gouvernement sur la question de la souveraineté numérique de la France, ou plutôt sur notre état de forte dépendance à l'égard de Google en matière d'agrégation de données. Je pourrais parler aussi de Palantir et de son actionnaire, la CIA, la DGSI y ayant eu recours pour gérer ses bases de données. L'expérience a démontré que l'échelle nationale ne permettra pas de résoudre ce problème et qu'il nous faut impérativement bâtir une stratégie d'indépendance informationnelle avec nos partenaires européens. Nous saluons la hausse des moyens consacrés à la mise en oeuvre de notre politique spatiale à l'échelle européenne. La recherche spatiale représentera en 2020 plus de 2 milliards d'euros. Ces crédits contribueront à apurer la dette de la France auprès de la France auprès de l'Agence spatiale européenne. Après le succès de la mission de Thomas Pesquet à bord de la station spatiale internationale et celui du GPS européen, Galileo, qui a dépassé le seuil du milliard d'utilisateurs cette année, nous assisterons, en juillet prochain, au vol inaugural du lanceur Ariane 6. La compétition La compétition mondiale s'accélère, s'exerçant au niveau tant des puissances étatiques que des acteurs privés. La Cour des comptes estime que notre politique spatiale manque encore d'ambition pour garder le cap face aux investissements massifs de la Chine et des États-Unis. Elle s'associe au Sénat pour appeler l'Europe à développer son propre lanceur réutilisable, à l'image de celui développé par SpaceX. Il serait illusoire de penser rivaliser avec les 21 milliards de dollars de budget annuel de la NASA, mais nous pouvons développer des points d'excellence dans des domaines précis, comme l'exploration des ondes gravitationnelles. Lors de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne réunie à Séville cette semaine, les vingt-deux pays membres ont voté une contribution globale de 14,3 milliards d'euros sur une période de trois à cinq ans pour intégrer la nouvelle donne internationale. Nous invitons le Gouvernement à positionner la France à la hauteur des enjeux auxquels l'Europe doit faire face. nous voterons les crédits de cette mission.

relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, mais aussi la réforme des études de santé et le plan Bienvenue en France, destiné à favoriser l'accueil des étudiants étrangers. étrangers. Permettez-moi de commencer par une remarque sur le contexte général dans lequel intervient ce budget. L'enseignement supérieur fait face depuis plusieurs années à une montée des effectifs liée au boom démographique de l'an 2000, dont on sait qu'il entraîne un accroissement automatique automatique du nombre d'étudiants. Le budget que vous présentez tient compte pour partie, pour partie seulement, de cette augmentation des effectifs. Il est certes en augmentation, ce que nous saluons, mais insuffisamment pour maintenir un budget par étudiant équivalent à celui de l'année dernière.

Espérons- ce n'est pas interdit ... -que, si l'État n'augmente pas mécaniquement le budget des universités quand les effectifs augmentent, il saura également ne pas le diminuer automatiquement quand les effectifs diminueront. diminueront. Les universités connaissent des tensions budgétaires d'autant plus fortes que l'accroissement des effectifs se cumule avec l'effet des réformes à mettre en place. Vous entamerez dans quelques jours une phase de dialogue avec les présidents d'université pour déterminer le montant de l'aide financière qui leur sera allouée. Nous avons compris que vous abordez cette phase avec une enveloppe de 50 millions d'euros à répartir et que la prise en compte du GVT ne sera pas automatique.

C'est pourquoi je formule d'ores et déjà la demande qu'un retour nous soit fait sur la répartition de cette enveloppe, une fois le dialogue de gestion terminé. aussi pour nous un moyen de comprendre les objectifs assignés par le ministère aux universités en matière de recrutement et d'accompagnement de leurs projets, pédagogiques ou de développement. De manière plus large, cela nous permettra également d'apprécier la pertinence et l'efficacité de cette phase de dialogue comme outil de pilotage. Les tensions budgétaires ont une autre conséquence, qui nous préoccupe tout particulièrement veux parler de l'état des bâtiments. Le parc universitaire est pour partie, s'agissant notamment des bâtiments construits dans les années 1970, vétuste et inadapté aux exigences environnementales. Il nécessite un effort financier de remise en état, sans même parler d'extension, un effort que les universités elles-mêmes ne peuvent fournir et que l'État, compte tenu de sa situation financière, ne peut supporter.

Par ailleurs, nous le savons, la réponse à la question immobilière repose en partie sur la dévolution aux universités elles-mêmes de leur patrimoine. Nous souhaitons connaître de manière précise le calendrier de ces dévolutions.

de la décision du Conseil constitutionnel, prise il y a quelques jours, sur les droits d'inscription. Elle pourrait inutilement mettre en difficulté les universités. Espérons que le Conseil d'État apportera une réponse rassurante sur ce sujet. Le budget pour 2020 est caractérisé aussi par la diminution du crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les donateurs aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Nous sommes

reflète la difficulté à disposer de données statistiques sur l'enseignement supérieur. De fait, l'outil statistique n'est malheureusement pas la hauteur de ce qu'il devrait être. Comparativement à d'autres ministères, par exemple celui de l'éducation nationale, nous sommes surpris de la faiblesse des données statistiques fournies sur l'enseignement supérieur. Résultat : il ne nous est pas possible d'apprécier les effets de certaines réformes que nous avons votées. Je pense en particulier au taux de réussite en première année de licence des étudiants, dont l'amélioration était pourtant l'un des objectifs majeurs de la loi Orientation et réussite des étudiants. Ces données nous sont essentielles pour savoir si les dispositifs d'accompagnement, les fameux « oui si », sont efficaces. Alors que nous sommes en période de discussion budgétaire, ces données éclaireraient fort utilement nos choix. Il nous serait également utile de savoir si l'effort indispensable d'augmentation des places en IUT et en BTS est mis en oeuvre et de connaître la part des bacheliers technologiques et professionnels en première année de ces filières. De même, et c'est une remarque plus personnelle, il serait intéressant de connaître l'impact de la mesure de régionalisation mise en oeuvre en Île-de-France cette année. Je voudrais maintenant aborder la question de la vie étudiante. L'événement dramatique de Lyon a placé dans le débat public la question du niveau des aides pour permettre la réussite des étudiants, mais aussi celle de la pertinence et de l'efficacité des dispositifs existants. Si nous sommes tous émus par ce geste dramatique, la réponse à ces questions ne saurait se limiter à la seule augmentation de lignes budgétaires. Elle suppose une analyse approfondie des dispositifs et des structures. Nous souhaitons vivement que cette analyse soit effectuée rapidement et sérieusement et que, à l'issue, des mesures soient prises pour aider les étudiants qui en ont besoin.

revalorisation indispensable de la fonction de chercheur par une rémunération tout simplement correcte, diversification nécessaire des financements, amélioration du lien entre recherche et développement industriel. Nous attendons les réponses du Gouvernement pour y faire face et leur transcription budgétaire. Il nous faudra pour cela attendre le projet de loi de finances pour 2021. Nous regrettons d'autant plus, dans ce contexte, la mesure d'augmentation du taux de réserve de précaution, qui nous paraît inappropriée au moment où la recherche devrait au contraire être aidée. Nous espérons, madame la ministre, que vous aurez gain de cause auprès de Bercy pour ne pas affaiblir inutilement nos outils en matière de recherche par un tour de passe-passe budgétaire dont le

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'augmentation de près de 1,7 % des crédits de la mission dont vous avez la charge a été saluée par tous les rapporteurs et presque tous les orateurs, cher Pierre Ouzoulias vous avez fait voter la loi Orientation et réussite des étudiants. Votre collègue Jean-Michel Blanquer avait lancé après vous, commettant une erreur manifeste de calendrier, la réforme du baccalauréat, dont je souhaite par ailleurs qu'il redevienne un tremplin pour la réussite des élèves dans l'enseignement supérieur. Assurément, votre volonté d'agir, comme celle de votre collègue de l'éducation nationale, demeure sincère et constante. Elle a été saluée. Reste la question des moyens. Ils sont en hausse, cela a été dit, et il faut vous en donner acte. Sont-ils pour autant suffisants compte tenu de l'impact des mesures déjà prises ? Sont-ils à la hauteur des défis de la recherche ? On sait que non, et les nuages menacent. C'est le cas, par exemple, du financement du glissement vieillesse-technicité, que vous semblez vouloir utiliser pour serrer la vis de certains. En 2018, il avait été intégralement compensé. En 2019, nous vous alertions sur l'utilisation d'une partie des crédits du plan Étudiants pour le financer. Pour 2020, vous avez annoncé que son financement ne sera pas systématique. Or la hausse globale peut masquer des situations très opposées, inscrites dans le temps long. Ainsi, le manque de moyens contraint certaines universités à ne pas remplacer les départs à la retraite, alors que nous devons répondre au défi que constitue l'arrivée de 30 000 étudiants supplémentaires chaque année. Autre motif d'alerte : depuis dix ans, sur le temps long, la dépense moyenne de l'État par étudiant stagne, voire diminue, masquant parfois des situations dramatiques. On le sait aussi, la vétusté des locaux s'aggrave, et la question de la précarité étudiante ne peut être passée sous silence. ce manque de financement de l'université ne date malheureusement pas d'hier, et on ne peut qu'acter l'effort réalisé cette année dans le cadre du projet de loi de finances. En revanche, l'abaissement du taux de défiscalisation des dons d'entreprises supérieurs à 2 millions d'euros marque un tournant. Limiter l'effet incitatif de ces dons risque de priver l'université de financements supplémentaires. On comprend mal pourquoi, dans ce contexte budgétaire difficile, vous affaiblissez le processus de diversification des sources de financement. Je partage donc pleinement l'alerte de notre rapporteur pour avis, Stéphane Piednoir, qui a pointé les conséquences de cette décision.

une refonte de la grille indemnitaire des chercheurs est nécessaire. C'est une question d'attractivité et de dignité. La baisse du nombre de doctorants doit faire l'effet d'un électrochoc. Permettez-moi, enfin, de vous interroger sur un point précis, majeur pour notre pays : la formation des professeurs du second degré, dont vous avez également la responsabilité en partage avec le ministre de l'éducation nationale dans le cadre des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. Ces instituts nationaux ont été maintenus au sein des universités, alors qu'ils auraient pu redevenir des écoles professionnelles intégrées au sein du ministère employeur. Je souhaite donc vous poser quatre questions. Comment les Inspé draineront-ils mieux que ne le faisaient les ÉSPÉ les ressources scientifiques de haut niveau que les élèves professeurs attendent et qui justifient l'ancrage des instituts de formation au sein de l'université ? Comment les maquettes de formation ne seraient-elles pas contraintes dès leur origine, comme le furent celles des ÉSPÉ, par les spécialités des enseignants qui y sont affectés ? Ce fut le point faible des défuntes écoles. Comment comptez-vous y remédier ? Comment les Inspé articuleront-ils mieux que ne le faisaient les ÉSPÉ la formation théorique et la formation pratique ? Comment s'établira la collaboration avec les corps d'inspection et les professeurs formateurs du second degré, sans que soit remise en cause l'autonomie des universités, mais de que les parcours des élèves professeurs soient rétablis en cohérence et en efficience ? C'était un point faible de la formation des ÉSPÉ. En conclusion, je voudrais réaffirmer que l'enseignement supérieur et la recherche ne pourront se passer d'une réforme profonde qui réponde durablement au défi de la démocratisation, de la compétition internationale et de la revalorisation du statut des chercheurs et des enseignants-chercheurs, au risque de voir notre pays poursuivre poursuivre son recul. Tel sera en particulier l'enjeu de la prochaine loi de programmation de la recherche. Dans cette attente, et au vu des efforts déjà déployés, comme les collègues de mon groupe, je voterai les crédits de cette mission.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant d'entamer l'examen proprement dit du budget, j'aimerais souligner le contexte très incertain qui l'entoure. En effet, par sa décision du 11 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a tiré du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 l'exigence constitutionnelle selon laquelle « la gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public ». Si des frais d'inscription « modiques » peuvent être perçus en tenant compte des « capacités financières des étudiants », il revient désormais au Conseil d'État de préciser la portée de ladite décision. Sur ce point, il convient de rappeler que la Cour des comptes, dans son rapport de novembre 2018, avait déjà alerté sur le développement de frais différenciés dans l'enseignement supérieur public, constatant un « écart croissant entre les modèles économiques des établissements » et soulignant le manque de cohérence du système. Quoi qu'il en soit, de la décision émanant des Sages, il paraît naturellement découler qu'un coût éloigné de l'exigence de gratuité représente une rupture réelle dans l'égal accès à l'instruction et ne saurait donc être constitutionnel. Ce contexte est d'autant plus source d'inquiétude pour les établissements du supérieur que leurs financements s'érodent, malgré les efforts que vous consentez, madame la ministre, puisque les crédits du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » augmentent d'un peu plus de 1 %. Néanmoins, cette hausse se révèle trop limitée, comme a alerté la conférence des présidents d'université après le vote à l'Assemblée nationale. Non seulement elle n'est pas de nature à couvrir la croissance démographique estudiantine- près de 33 000 étudiants supplémentaires se sont inscrits à la rentrée de 2019 et près de 15 000 nouveaux étudiants sont attendus en 2020 mais elle ne permet pas non plus de mettre en oeuvre correctement les multiples réformes engagées : la loi ORE, la loi pour une école de la confiance, qui pose la question essentielle du continuum entre le lycée et l'enseignement supérieur, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, bien sûr, la réforme des études de santé. Au final, les universités ont chiffré à 250 millions d'euros les moyens financiers complémentaires nécessaires. Or, en valeur réelle, le budget qui leur est alloué ne croît « que » de 160 millions d'euros, soit un écart de 90 millions d'euros forcément préjudiciable. Ce problème de financement chronique se double aujourd'hui d'une pression accrue sur les ressources propres des établissements, créant ainsi un véritable effet ciseau qui risque d'avoir des conséquences désastreuses sur leurs investissements en faveur des étudiants ou de la rénovation énergétique des bâtiments.

qui, sans aucun doute, aboutira à un effet d'éviction. En outre, elle portera un coup à l'intensification des partenariats entre les établissements du supérieur et les acteurs économiques, qui participent pourtant de la structuration territoriale. C'est pourquoi notre commission proposera de maintenir le régime prévalant pour le mécénat.

À travers ces différentes difficultés est profondément posée la problématique du financement de l'enseignement supérieur. Outre la solidité et la soutenabilité financières des universités, l'enjeu sous-jacent est bel et bien celui de la réussite des étudiants au sein de formations qualifiantes et, par là même, de la capacité de la France à innover et à rayonner. Nous ne pouvons nous résoudre à ce que le financement par étudiant inscrit à l'université ait atteint son plus bas niveau depuis dix ans, plafonnant à un peu plus de 10 000 euros et, surtout, accusant une baisse de plus de 1 000 euros en quelques années seulement. Nous avons collectivement un devoir envers la jeunesse : lui assurer un avenir malgré les défis colossaux qui l'attendent. Cet avenir passe obligatoirement par une formation de qualité tout au long de la vie,

inflation générale du coût de la vie, qui oblige certains à subir un emploi à temps partiel, renoncement aux soins, loyer onéreux, etc. Si nous ne pouvons que saluer l'accroissement de 46 millions du montant alloué aux bourses sur critères sociaux ainsi que la récente décision de geler les loyers des résidences universitaires, l'effort budgétaire ne nous paraît pas à la hauteur de la situation. Nous présenterons un amendement visant à réinjecter les 35 millions d'euros que le Gouvernement a gelés sur le programme « Vie étudiante » en 2019. En outre, nous appelons à accélérer les réflexions en cours pour créer une allocation d'autonomie à destination de tous les étudiants en situation de précarité. Sans remettre en cause l'absolue nécessité des bourses sur critères sociaux, il paraît fondamental de gommer l'effet de seuil excluant des jeunes qui devraient légitimement bénéficier d'une aide financière de l'État. Autrement dit, nous ne souhaitons pas uniquement une revalorisation des bourses : nous voulons un changement systémique et d'échelle, une vraie réforme. Madame la ministre, y êtes-vous prête ? ? Les discussions actuelles vont-elles dans ce sens ? En ce qui concerne le budget affecté à la recherche, le contexte est quelque peu particulier, puisque, mes collègues l'ont dit, la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche est annoncée pour le début de l'année prochaine et que beaucoup de réponses à nos interrogations sembleraient devoir s'y trouver. Par conséquent, nous espérons qu'elle sera à la hauteur des nombreuses attentes et ambitions affichées. Pour l'instant, force est de constater que les moyens dévolus dans le cadre de ce PLF n'enthousiasment pas le monde de la recherche. En cause, singulièrement, la stagnation du crédit du programme 172 relatif à la recherche pluridisciplinaire, qui concentre les principaux opérateurs nationaux. En parallèle, le taux de réserve appliqué aux instituts demeure assez élevé, tout particulièrement pour l'ANR. En 2019, celui-ci s'est élevé à 8

pouvez-vous nous préciser le taux de réserve que vous entendez appliquer en 2020 ? S'agissant de l'intelligence artificielle, thématique d'avenir par excellence, nous nous réjouissons que le plan national lancé en 2018, trouve sa traduction budgétaire au sein du Érigé au rang de priorité par la Commission européenne, l'investissement en la matière doit favoriser le rattrapage de l'Europe sur les États-Unis et la Chine. Si le retard accumulé depuis vingt ans est important, je ne pense pas qu'il soit insurmontable à une double condition avoir un environnement économique et scientifique favorable à l'innovation et coordonner les actions des États membres pour ne pas tomber dans l'écueil d'une compétition intra-européenne qui ne peut conduire qu'à un résultat perdant-perdant. L'accent mis sur l'IA doit impérativement aller de pair avec l'affirmation d'un État de droit numérique. L'accélération des progrès technologiques ne peut se faire en dehors de tout cadre démocratique, comme si, finalement, les avantages tirés des nouvelles applications pouvaient justifier des atteintes croissantes et disproportionnées aux libertés publiques. Tout ne peut être permis. L'Europe doit faire émerger encore plus rapidement son modèle pour mieux protéger ses citoyens. En cela, le RGPD constitue une première pierre vraiment importante de l'édifice, qui doit être encore consolidé, car, comme il a été démontré dans un récent rapport sénatorial, en filigrane se jouent à la fois notre souveraineté et la souveraineté numérique de l'Europe, ainsi que la création et la captation de richesses par le truchement des données personnelles notamment.

En France, leur précarisation, en particulier en début de carrière, est réelle. Il s'ensuit mécaniquement une perte d'attractivité, comme le prouve la diminution du nombre de doctorants. nombre de doctorants. Dans la perspective de la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, nous espérons vraiment que le Gouvernement s'attachera à améliorer le traitement des chercheurs. Nous y serons extrêmement vigilants. Madame la ministre, mes chers collègues, au regard de toutes les inquiétudes et de toutes les réserves exprimées, et en l'état, il s'avère impossible pour nous de voter les crédits de cette mission, mais nous espérons que la future loi de programmation lèvera demain

concernant la progression des crédits alloués à la recherche, malgré les réserves émises par nos rapporteurs, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Comme il faut choisir ses thèmes, je commencerai par la première priorité en volume financier notre politique spatiale, qui relève d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres depuis l'adoption du traité de Lisbonne. Les 214 millions d'euros supplémentaires sont destinés à apurer la dette française à l'égard de l'Agence spatiale européenne, ce qui permet à la France de crédibiliser son engagement dans les programmes spatiaux européens. Plus qu'une obligation, c'était une nécessité ! Vous le savez, le Parlement s'est beaucoup investi dans la préparation des enjeux de la conférence de Séville, dont vous revenez. L'Opecst travaille depuis longtemps sur ces sujets.

J'espère que vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus. L'année 2020 nous permettra de savoir si les choix technologiques et budgétaires pour le futur lanceur Ariane 6 ont été les bons. Mais, nous le savons tous, son succès commercial dépend aussi de l'engagement des pays contributeurs à lui confier leurs lancements institutionnels. Malheureusement, je n'ai pas vraiment l'impression que cela progresse. La recherche spatiale, ce ne sont pas que les lanceurs, ce sont aussi les satellites. Sans eux, les prouesses de nos fusées ne seraient qu'une réussite scientifique coûteuse.

Mais qu'en est-il des services payants qui devaient rentabiliser Galileo ? Cette année, je passerai brièvement sur l'ANR. Grâce aux moyens financiers supplémentaires qui lui sont alloués en 2020, elle pourrait sélectionner 800 projets supplémentaires par rapport à 2018, où ils où ils furent près de 1 500. Mais, avec un taux de sélection de 16,2 %, nous sommes encore loin de la moyenne des pays européens, qui est de 25 %, ni surtout de la simplicité pour concourir. Avec un taux d'échec de 85 % des projets présentés, la démotivation des équipes est légitime eu égard à l'effort administratif et à la complexité que demande le dépôt d'un dossier. J'espère, madame la ministre, que vous n'allez pas donner un poids démesuré à l'ANR dans votre prochaine loi de programmation, car vous risqueriez de décourager les chercheurs. Il faut les écouter quand ils demandent une amélioration du fonctionnement de l'Agence en matière de transparence et une meilleure adaptation à chacune des disciplines scientifiques. En matière de recherche sur l'énergie nucléaire, nous sommes nombreux, en tout cas au sein de l'Opecst, à être soulagés concernant le réacteur expérimental Jules Horowitz, que j'appellerai RJH. À une période où l'on s'interroge sur la durée de vie de nos centrales actuelles, sur la fiabilité des équipements et où l'on espère enfin voir fonctionner l'EPR retardé par la fiabilité de soudures et de tuyauteries, l'utilité de ce réacteur expérimental est encore plus évidente. Rappelons qu'il fournira des données scientifiques sur le comportement des composants et des combustibles nucléaires. L'impasse financière devant laquelle se trouvait le CEA pour finir la construction du RJH n'était pas acceptable. En revanche, il ne produira pas d'énergie, contrairement aux réacteurs de quatrième génération. L'abandon du réacteur à neutrons rapides Astrid, qui aurait permis de recycler à l'infini le combustible nucléaire, est à mes yeux une erreur scientifique. scientifique. Ce n'est pas une décision politique qui en est l'origine, mais une raison économique, selon l'administrateur du CEA, qui a déclaré devant la commission des affaires économiques que l'uranium n'était plus assez cher pour justifier des dépenses pour le recycler, même en produisant de l'électricité.

Décidément, l'histoire bégaie en matière de recherche nucléaire sur les réacteurs de nouvelle génération, et je le regrette. Pour terminer mon propos, j'évoquerai le CIR, qui est un outil indispensable au développement de la recherche. L'État se doit d'encourager les entreprises à investir en R&D, source d'innovation et d'attractivité. Si certains s'interrogent sur l'efficacité du CIR

d'argent public reçu. Le CIR a permis de redresser l'effort de la France en R&D. Dans notre pays, où la fiscalité des entreprises est au plus haut, évitons que celles-ci ne partent ailleurs en Europe. je salue l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale, qui est revenu sur l'obligation documentaire instaurée l'an dernier par les députés. Il faudra veiller, dans votre future loi de programmation, à ne pas déshabiller Paul pour habiller Pierre.

Les mesures et les moyens du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », dont le champ couvre l'ensemble des fonctionnaires de l'État, ne sont pas complètement adaptés à la situation des chercheurs, particulièrement à la situation des chercheurs ayant effectué un beaucoup de difficultés à retrouver un poste en France. Une étude portant sur 400 jeunes chercheurs français partis après leur doctorat entre 2003 et 2008 a montré que 57 % d'entre eux résidaient encore à l'étranger

Monsieur le président, messieurs les rapporteurs spéciaux, madame, messieurs les rapporteurs pour avis, avis, mesdames, messieurs les sénateurs, l'examen des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » est, comme chaque année, un rendez-vous qui doit nous permettre d'évoquer l'ensemble des sujets qui relient l'enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. C'est un temps important pour le Parlement, tout particulièrement pour le Sénat, mais c'est également un moment très attendu par l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur. D'emblée, D'emblée, au nom du Gouvernement, je tiens à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, dans nos universités, nos écoles, nos laboratoires de recherche et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires, font vivre au quotidien cette exigence qui est au coeur de la mission qui sera soumise à vos suffrages dans quelques instants. Si ce rendez-vous est chaque année si important pour la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, il revêt aujourd'hui un caractère particulier, chacun a pu le mesurer dans cet hémicycle. Le drame survenu le 8 novembre dernier à Lyon a jeté une lumière sans fard sur les conditions de vie de certains étudiants confrontés à des situations de précarité sans avoir connaissance des dispositifs qui peuvent les aider au quotidien. Améliorer les conditions de vie des étudiants est une priorité de mon ministère. Plusieurs réponses sont d'ores et déjà apportées par le projet de budget pour 2020. J'y reviendrai. Si la jeunesse est au coeur des politiques conduites par mon ministère, c'est que le champ de la Mires est intégralement dédié à préparer l'avenir de notre nation. Former notre jeunesse, construire un agenda de la connaissance scientifique au service du rayonnement de la France

C'est parce que le Gouvernement a pleinement conscience de cet enjeu pour notre avenir que la Mires fait partie des missions prioritaires du prochain budget triennal. S'agissant de l'année 2020, le budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, tel qu'il a été présenté par le Gouvernement, est composé de 25,35 milliards d'euros en crédits de paiement. Avec une hausse de 500 millions d'euros par rapport à 2019, la Mires a fait l'objet d'un effort considérable de la part du Gouvernement, un effort qui représente à lui seul 10 % des crédits nouveaux de l'État. Naturellement, ces sommes déjà considérables ne représentent pas à elles seules l'effort général de la Nation envers notre jeunesse et notre recherche. À ces 25,35 milliards d'euros s'ajouteront les 140 millions d'euros de recettes de la contribution de vie étudiante et de campus versées directement aux établissements d'enseignement supérieur et aux Crous. Le programme d'investissements d'avenir joue par ailleurs, comme vous le savez, depuis plus d'une dizaine d'années, un rôle majeur dans la recomposition du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Enfin, les collectivités territoriales jouent un rôle chaque jour plus important en matière de financement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Certains d'entre vous ont joué un rôle pionnier en la matière. Je songe naturellement au travail considérable que vous avez réalisé, monsieur le sénateur Adnot, pour la création de l'université technologique de Troyes. Cet engagement des collectivités n'est à mon sens pas encore assez reconnu. Je gage que votre rapport, monsieur le sénateur Rapin, permettra de mieux faire connaître cet effort cet effort significatif et important. Comme cela a été évoqué par plusieurs intervenants, l'année 2020 sera avant tout consacrée à la préparation et à l'examen du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, annoncé en février dernier par le Premier ministre et confirmé cette semaine par le Président de la République.

Une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche est un événement rare. Le Président de la République comme le Premier ministre ont exprimé le souhait que cette programmation pluriannuelle puisse débuter dès le début de l'année 2021, c'est-à-dire dans le cadre d'un calendrier harmonisé et mis en cohérence

mais également avec celui du programme Horizon Europe, qui, comme vous l'avez rappelé, sera le programme de recherche le plus ambitieux jamais élaboré. Vous l'aurez compris, l'un des enjeux de la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche sera de mieux articuler les politiques régionales, les politiques territoriales et nationales de l'État et la capacité de nos chercheurs à faire valoir l'originalité de leurs travaux à l'échelon européen. À cette fin, le budget pour 2020, dernier budget avant cette loi de programmation, permettra de soutenir et d'amplifier toutes les initiatives d'ores et déjà lancées par mon ministère depuis le mois de mai 2017. Comme vous le savez, et c'est une conviction que je rappelle chaque année, il ne faut pas opposer le soutien non thématisé à la recherche et le soutien à des sujets spécifiques. Ce projet de loi de finances permettra d'augmenter de 32,7 millions d'euros par rapport à l'an dernier les moyens d'engagements de l'ANR. Le plan Intelligence artificielle montera en puissance, passant de 17 millions à 38 millions d'euros dès 2020, soit une augmentation de plus de 100 %.

la mesure de soutien à la coordination en matière de recherche fondamentale dédiée à la lutte contre les cancers pédiatriques. Ce sont 5 millions d'euros qui seront dédiés à ce dispositif en complément des programmes d'ores et déjà pilotés et financés par l'INCa et l'Inserm. Le climat et le développement durable sont également des priorités affirmées par mon ministère et ont fait l'objet de deux programmes prioritaires de recherche. Je songe évidemment au programme Mopga et à celui consacré à l'agriculture. Au-delà, l'investissement dans les programmes spatiaux, notamment les programmes d'observation de la Terre, ainsi que le succès de la conférence ministérielle de l'ESA nous permettent d'affirmer que le climat et la surveillance du climat font partie des priorités, non seulement de la France, mais aussi de l'Europe. Le succès de cette conférence ministérielle doit d'ailleurs beaucoup à l'unité dont ont fait preuve le Gouvernement et les parlementaires, notamment les sénateurs, pour soutenir l'excellence de la recherche et de l'industrie françaises. Dans le cadre de la fusion entre l'INRA et l'Irstea, mon ministère accompagnera la création de l'Inrae, grâce à une dotation de 2,5 millions d'euros supplémentaires. Ce nouvel organisme organisera et coordonnera tous les travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la gestion durable des territoires et de la prévention des risques. Tous les chercheurs ont en commun une vocation chevillée au corps et dédiée à l'exploration de la connaissance. Cette vocation, que je partage avec certains d'entre vous, rend d'autant plus criante la question de la rémunération des chercheurs et des enseignants-chercheurs. En attendant les mesures qui seront prises en ce sens dans la loi de programmation, nous portons une attention particulière à l'emploi et à l'attractivité des carrières scientifiques dans ce budget, notamment au sein des organismes de recherche. Près de 28 millions d'euros seront consacrés aux PPCR Ce budget permettra ainsi de soutenir la politique de ressources humaines des organismes de recherche. Près de 12 millions d'euros supplémentaires seront en outre consacrés au CNRS, qui, par ailleurs, déploiera dès 2020 un pack d'accueil d'un montant moyen de 10 000 euros pour ses nouveaux chargés de recherche d'une enveloppe budgétaire de 2,5 millions d'euros. Le soutien à l'équipement et aux infrastructures est également fondamental pour l'année à venir. Dans le domaine spatial, 226 millions d'euros supplémentaires serviront à tenir nos engagements auprès de l'ESA et près de 15 millions d'euros de plus contribueront à soutenir les activités du CNES. À l'occasion de la conférence ministérielle de Séville, j'ai eu à coeur de défendre le leadership européen de notre pays en matière spatiale. Des engagements forts ont été pris par la France en la matière. que ministre chargée de l'espace, j'aurai l'occasion d'en rendre compte devant la commission des affaires étrangères et de la défense ainsi que devant la commission des affaires économiques, qui ont souhaité, dans un récent rapport d'information, s'emparer de la question des lanceurs.

Les universités, c'est l'une de leurs principales missions, jouent un rôle à part entière d'opérateurs territoriaux de la recherche en lien avec leurs missions de formation et d'insertion professionnelles au service de notre jeunesse. Je souhaite naturellement que cette vocation historique des universités sorte renforcée de la loi de programmation et que chaque université puisse y trouver les outils pour affermir sa signature. Dans l'immédiat, le budget pour 2020 permettra de poursuivre le déploiement du plan Étudiants et de financer toutes les missions des universités. Le programme 150 verra ainsi ses crédits augmenter de 176 millions d'euros. La trajectoire fixée dans le projet de loi de finances pour 2018 sera belle et bien respectée. Depuis 2017, ce sont 542 millions d'euros supplémentaires qui sont venus consolider le budget du programme 150, sans compter la contribution du programme d'investissements d'avenir à hauteur de 350 millions d'euros, qui sont alloués à la réforme du premier cycle. cycle. Près de 142,5 millions d'euros seront consacrés au plan Étudiants, soit 43 millions d'euros de plus que l'an passé. Ces moyens permettront à nos universités d'ouvrir des places supplémentaires et d'approfondir les dispositifs de remédiation mis en place par la loi Orientation et réussite des étudiants. Derrière les chiffres et les statistiques, ce qui se joue actuellement dans les universités, c'est la confirmation d'un changement qui est à l'oeuvre depuis l'année dernière grâce à Parcoursup, à la nouvelle politique d'orientation, pour laquelle je tiens à à remercier l'ensemble des enseignants du secondaire et l'ensemble des services responsables de l'orientation qui y contribuent, ainsi qu'au phénomène de remédiation. Pour ne prendre qu'un seul exemple, en Staps, le taux de réussite a progressé de 11,7 points en un an. Des évaluations sont en cours, et j'aurai à coeur de rendre compte devant vous des effets du plan Étudiants sur la réussite des étudiants en licence lors d'une audition prévue en début d'année Outre la mise en oeuvre du plan Étudiants, deux autres transformations structurelles sont à l'oeuvre dans l'enseignement supérieur. Tout d'abord, nous généralisons en 2020 le dialogue stratégique et de gestion avec les établissements, qui doit nous permettre de rénover en profondeur les modalités d'allocation des moyens versés aux universités. Ce dialogue permettra de répartir une enveloppe de 50 millions d'euros. Une autre enveloppe de 50 millions d'euros sera directement affectée au financement du PPCR pour 2020, ainsi qu'à la reconnaissance de l'investissement pédagogique. Naturellement, j'entends vos analyses, monsieur le rapporteur spécial Adnot. Après l'expérimentation conduite l'année dernière sur treize établissements, nous franchissons une deuxième étape en généralisant la démarche sur l'ensemble du territoire. Une fois que le dialogue stratégique sera effectivement lancé et appliqué, viendra le temps de son approfondissement. L'enjeu pour l'année à venir est de fournir à l'État un levier pour ouvrir une discussion globale avec les établissements sur leur gestion annuelle, leurs charges, leurs ressources, mais surtout sur leurs projets et leurs réels besoins d'accompagnement. C'est bel et bien à ce niveau que se situe l'originalité du dialogue stratégique et de gestion. Autre transformation majeure : la réforme des études de santé. Sur le plan budgétaire, plus de 16 millions d'euros supplémentaires seront versés pour soutenir les initiatives pédagogiques et innovantes dans les établissements. S'agissant de la vie étudiante, sujet au coeur des préoccupations du Gouvernement, comme je l'ai rappelé au début de mon intervention, et dans le contexte tragique que chacun connaît ici, ici, je tiens à rappeler que près de 5,7 milliards d'euros sont annuellement consacrés, la Mires, les aides au logement ou la protection sociale, à l'effort de solidarité de la Nation envers nos étudiants. Je ne crois pas me tromper en affirmant que peu de pays dans le monde sont capables d'afficher un tel effort continu et croissant depuis plusieurs décennies. Cette année, les moyens budgétaires du programme 231 sont en hausse de 67 millions d'euros. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous avons revalorisé les bourses sur critères sociaux. Naturellement, le Gouvernement reste à l'écoute des revendications qui s'expriment, afin de faire face aux situations de grande précarité traversées par de nombreux étudiants. Pour y remédier, j'ai d'ores et déjà pris plusieurs mesures d'urgence. Dès le 20 novembre dernier, j'ai demandé au réseau des oeuvres universitaires et scolaires d'appliquer la trêve hivernale au bénéfice de tous les étudiants en difficulté qui résident dans une résidence du Crous. Pour tous, il a été décidé de geler les loyers, ce qui représente un effort financier de 6 millions d'euros environ, qui sera réalisé en gestion. Pour les situations les plus difficiles, il existe des dispositifs qui sont d'ores et déjà financés, mais souvent trop peu et trop mal utilisés. Je songe notamment aux aides d'urgence, qui peuvent aider à tout moment de l'année les étudiants les plus en difficulté à sortir d'une situation de grande précarité. Nous savons que de nombreux étudiants subissent au quotidien des problèmes importants sans savoir où s'adresser ou sans oser faire appel au réseau des oeuvres. année, ce sont plus de 15 millions d'euros d'aides qui ne sont pas consommés. Nous avons l'obligation de faire mieux. Aussi, je souhaite qu'un véritable fonds consacré aux aides d'urgence soit instauré et que tous les moyens soient mis en oeuvre pour le faire connaître, les Crous, les établissements d'enseignement supérieur et les associations étudiantes. Un numéro vert sera aussi mis en place à cette fin. Ces mesures s'inscrivent dans le prolongement du travail réalisé par le ministère pour améliorer les conditions de vie des étudiants et des boursiers. Je pense évidemment à la suppression de l'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants, généralisée à l'ensemble des étudiants depuis la rentrée de septembre. Près de 200 millions d'euros sont dorénavant pris en charge par la sécurité sociale au profit de la santé de nos étudiants. Je songe également à la mise en oeuvre de la contribution de vie étudiante et de campus, qui devrait générer cette année et l'an prochain près de 140 millions d'euros, notamment consacrés au financement d'actions de prévention sanitaire et d'action culturelle. À cet égard, il a été décidé, conjointement avec la CPU, que la santé physique et psychologique des étudiants serait la priorité principale de l'emploi de la CVEC en 2020. Naturellement, madame la sénatrice Robert, le régime même des bourses sur critères sociaux doit être substantiellement révisé. C'est un débat que le Sénat a souhaité ouvrir à l'occasion de la loi Orientation et réussite des étudiants en évoquant la question de l'assiduité des étudiants, dans le prolongement de vos travaux, monsieur Adnot.

qui, souvent, évincent de trop nombreux étudiants. Voilà en quelques mots et en quelques minutes les principales lignes de force de ce budget pour 2020. J'aurai l'occasion d'apporter d'autres précisions lors de l'examen des amendements. d'un budget sincère, d'un budget prioritaire, construit en responsabilité, et c'est ce budget que le Gouvernement vous propose d'adopter. Nous allons

Notre rapporteur spécial estime, et je partage complètement son avis, qu'il serait nécessaire de doter l'ANR d'un budget d'environ 1 milliard d'euros, ce qui me semble être une estimation tout à fait valable.

Vous le savez aussi, la moitié des étudiants travaillent à mi-temps pour payer leurs études. Pour avoir enseigné à l'université, je peux vous assurer que l'on ne peut pas faire de bonnes études quand on livre des pizzas une partie de la nuit.

notamment dans les métropoles, où les prix de l'immobilier s'envolent et où il devient de plus en plus difficile pour les étudiants de se loger. L'Observatoire national de la vie étudiante devrait rendre un rapport

afin de discuter ensemble de la précarité étudiante et des moyens que nous pourrions mettre en oeuvre pour y remédier. Quel est

pour que cet outil reprenne tout son sens. C'est ce qui est fait, projet de loi de finances après projet de loi de finances, et c'est évidemment un sujet qui sera abordé dans la loi de programmation pour la recherche.

auprès des régions, parce qu'ils considèrent que, pour un chercheur en sciences humaines, l'ANR est devenu un guichet trop difficile d'accès.

et indispensables pour aider les start-up, les TPE et les PME dans les phases les plus risquées de leur développement, lorsqu'elles ne bénéficient pas encore de la solidité suffisante pour obtenir un soutien bancaire privé. La France connaît depuis le début des années 2010 un vrai développement économique l'innovation. Le nombre de nos start-up ne cesse de croître, notamment grâce à l'impulsion d'acteurs publics en faveur de l'innovation des entreprises. C'est le cas de Bpifrance, qui finance des projets innovants, principalement sous la forme d'aides individuelles directes aux entreprises, et notamment les PME innovantes. Ces aides sont majoritairement financées par l'État sur le programme 192, qui joue un rôle bien plus important que le Fonds pour l'innovation et l'industrie, dont personne ne comprend véritablement la vocation. J'ajoute que ces crédits ont la particularité d'accompagner de nombreux projets au coeur de nos territoires, dans toutes les régions, et pas seulement dans des zones denses des métropoles. Ils ont donc un intérêt particulier en termes d'aménagement du territoire. Après un abondement de 250 millions d'euros en 2011, les moyens de l'État gérés par Bpifrance ont

alors même que le rapport sur les aides à l'innovation, élaboré par Jacques Lewiner, Ronan Stephan, Stéphane Distinguin et Julien Dubertret, et remis au Gouvernement en mars 2018, préconise de maintenir les aides à l'innovation de Bpifrance inscrites dans le programme 192 à un niveau de 140 millions d'euros minimum.

le rapporteur pour avis. Avec cet amendement, la commission des affaires économiques souhaite interpeller le Gouvernement sur la cohérence de sa politique en faveur de l'innovation. Nous sommes bien conscients de l'effort financier réalisé en faveur de la recherche et de l'innovation, mais l'enveloppe des aides à l'innovation, qui reste modeste, devrait être sanctuarisée. L'effort demandé au Gouvernement est limité. Notre commission avait alerté l'année dernière sur la nécessité de ne pas descendre en dessous de 120 millions d'euros de dotations finançant les aides à l'innovation de Bpifrance. Nous étions déjà indulgents, car le rapport sur les aides à l'innovation plaidait pour ne pas descendre en deçà de 140 millions d'euros. le Gouvernement propose de nouveau de diminuer cette dotation, qui chuterait à 100 millions d'euros. Les politiques d'innovation doivent être claires et stables, sans quoi elles s'apparentent à de véritables coups d'épée dans l'eau. Madame la ministre, vous nous direz probablement que le Fonds pour l'innovation et l'industrie compense cette baisse des crédits. Mais, d'une part, nous n'apprécions pas ce fonds, car il nous prive de notre droit de regard annuel sur 250 millions d'euros et, d'autre part, vous savez que la cible du plan Deep Tech n'est pas la même que celle des aides à l'innovation. Dans un cas, il s'agit de financer l'innovation à la sortie du laboratoire ; dans l'autre, il s'agit de financer toutes les entreprises innovantes de notre territoire. Pourquoi se priver d'un tel instrument dont l'effet de levier est majeur ? Il irrigue toutes les entreprises de notre territoire, et il a prouvé son efficacité, tant au regard de la croissance des entreprises concernées que du taux élevé de remboursement des aides. Madame la ministre,

Notre rapporteur spécial Philippe Adnot a rappelé, très justement, que le Gouvernement s'était engagé en 2017 à construire 60 000 logements et qu'il y a peu d'espoir que la moitié de ces logements soient réellement livrés avant la fin de la mandature.

les objectifs fixés sont absolument inatteignables. En revanche, vous venez d'annoncer, madame la ministre, le gel des loyers pour la totalité du parc des résidents du Crous. Bien évidemment, on ne peut être que très favorable à cette mesure, qui sera prise en charge intégralement par votre ministère, à hauteur de de 6 millions d'euros. Néanmoins, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2019, le Gouvernement a proposé, et obtenu, la suppression de près de 35 millions d'euros de crédits destinés à la vie étudiante. Je vous rappelle que ce montant correspond à des crédits entièrement gelés en début d'exercice et, ensuite, totalement annulés. La loi de finances rectificative a été définitivement adoptée par le Parlement le 26 novembre. Trois jours après,

destiné aux aides directes aux étudiants, que le Gouvernement supprimait. Malheureusement, le rétablissement de ces crédits n'a pas survécu à l'examen en CMP du PLFR pour

35 millions d'euros supplémentaires ne seront pas superflus pour renflouer les bourses, dont seul le taux sera réévalué de 1,1 % en 2020, après quatre exercices de stagnation et, donc, de baisse en valeur constante, pour accroître les aides au mérite, qui accusent en 2020 une chute pour la deuxième année consécutive, pour amplifier les aides à la mobilité internationale et aux mobilités Parcoursup ou master. Alors que la précarité étudiante grandissante a été révélée à l'occasion du geste dramatique d'un jeune, il n'est pas responsable de poursuivre les coupes budgétaires dans les crédits de l'année en cours, crédits destinés à contribuer à remédier à ces conditions de vie et d'études déplorables.

pas en métropole. Je rappelle que la précarité étudiante en outre-mer est supérieure de 7 points à celle des étudiants de l'Hexagone

favoriser le développement d'une capacité nationale d'innovation, dont les résultats seront utilisables par l'ensemble des acteurs du secteur, et,, garantir aux consommateurs une alimentation saine, sûre et accessible à tous. Cette proposition consacre une préconisation formulée dans le cadre des États généraux de l'alimentation, qui suggérait la mise en place d'un dispositif de soutien des instituts techniques agro-industriels. L'amendement tend donc à diminuer les crédits des actions n 11 et 12 du programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

de l'enseignement supérieur et de la recherche agricoles. Dans le contexte actuel, où il est nécessaire d'engager des recherches fortes pour permettre une mutation

Le concept de la « santé personnalisée » est introduit comme objectif prioritaire de la politique nationale de santé et de la politique publique de recherche et d'innovation. Afin d'en accompagner le développement, il est proposé de flécher les financements de la recherche vers les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère industriel et commercial et d'autres opérateurs publics intervenant dans la recherche et développement ou l'innovation en matière de santé personnalisée. Mme Berthet tend à créer un nouveau programme au sein de la mission « Recherche et enseignement supérieur », intitulé « Recherche scientifique et technologique pour la santé personnalisée », en retirant 10 millions d'euros à l'action n° 03, Recherche culturelle et culture scientifique. Si toutefois il y avait une demande de retrait,

un nom aux racines historiques pour le distinguer de la recherche publique et de la recherche privée, comme on distinguait le tiers état de la noblesse et du clergé. Depuis les années 1970, en écho à l'émergence dans la sphère publique de diverses controverses sanitaires, environnementales ou sociétales, plusieurs secteurs de la société civile se sont mobilisés, afin de développer leur propre capacité d'analyse, de réflexion et d'action, constituant une expertise citoyenne en contrepoint de l'expertise scientifique officielle, souvent suspectée de ne pas éclaircir correctement les enjeux d'un certain nombre de décisions publiques. Quarante ans plus tard, la mobilisation de cette expertise citoyenne s'est considérablement développée dans les territoires, d'un secteur dénommé « tiers secteur de la recherche », qui regroupe des acteurs divers- entreprises, associations, élus locaux -associés dans des formules en réseau très variées. Ce secteur présente aujourd'hui une réelle capacité à faire émerger des champs et des thématiques de recherche innovants et des solutions adaptées à des sujets peu pris en compte par la recherche publique ou privée, sujets que l'on peut qualifier d'orphelins. peut qualifier d'orphelins. Il tend à donner un souffle nouveau à l'innovation, notamment dans le champ du numérique et de l'écologie. Il produit des segments de recherche et développement partant du terrain et des expertises associatives et entrepreneuriales en plein développement. L'objet du présent amendement est de faire reconnaître officiellement cette approche et que ces tiers lieux puissent bénéficier, pour partie, de prérogatives comparables à celles des laboratoires de recherche traditionnelle, en termes de recours aux dispositifs financiers ou de soutien à la recherche. et c'est là que le bât blesse, de financer un programme « Tiers secteur de la recherche » par un abondement de 8,5 millions d'euros prélevés sur les actions n 11 et 12 du programme 172.

travaillent de façon tout à fait bénévole ! On parle beaucoup du taux d'abandon des études en licence. Le taux d'abandon en doctorat est aussi

de crédits de l'action n° 14, Immobilier, du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », vers l'action n° 01, Aides directes, du programme 231 « Vie étudiante Cette somme correspond au montant que coûterait l'octroi de bourses aux étudiants calédoniens qui ont vu leur demande refusée, en raison de l'inadaptation des plafonds d'éligibilité « métropolitains » à la vie particulièrement chère en Nouvelle-Calédonie.

En abondant les crédits des bourses sur critères sociaux, l'État rend possible la proposition d'une modulation des critères d'éligibilité pour les territoires spécifiques de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie, afin que les enfants issus des familles modestes ne soient pas privés de la chance de poursuivre un cursus dans l'enseignement supérieur.

la séance et la commission de leur mansuétude, qui me permet d'évoquer le problème des droits d'inscription à la suite de la récente décision du Conseil constitutionnel. La séance m'a proposé de déposer un rapport,

et d'une contribution supplémentaire au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le réacteur universitaire de Strasbourg n'est plus exploité depuis

a présenté plusieurs mesures visant à améliorer la compétitivité et l'attractivité de la France dans le domaine de la santé, notamment dans la recherche et le développement des biomédicaments et des thérapies innovantes. Ces mesures visent notamment à permettre le développement d'une filière de médicaments de thérapie innovante.